La séance est ouverte..

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique est parvenue à l'adoption d'un texte commun. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la prescription en matière pénale et du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse,

M. Le président du Sénat a reçu de M. le président de l'Assemblée de la Polynésie Française, par lettre en date du 26 janvier 2017, les rapports et les avis sur -le projet d'ordonnance modifiant la partie législative du code des juridictions financières ; -le projet d'ordonnance prise en application de l'article 216 de la loi n° 2016 41 du 26 janvier 2016 et relatif à la lutte contre la propagation internationale des maladies ; -et le projet d'ordonnance relatif à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la réglementation de l'alcoolémie en mer. Acte est donné de ces communications. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales,

Les échanges que nous avons eus ici et à l'Assemblée nationale ont déjà été longs, riches, souvent fructueux- je m'en félicite -et parfois vifs- je m'en étonne, je ne vous le cache pas. J'étais certaine que, plus de quarante ans après son adoption, la loi Veil faisait aujourd'hui largement consensus. Le texte que vous allez de nouveau examiner visait d'ailleurs non pas à rouvrir le débat sur l'avortement, mais simplement à permettre à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes d'exercer cette liberté de disposer de leur corps. En proposant d'étendre le délit d'entrave à l'IVG au monde numérique, vos collègues députés n'avaient pas d'autre ambition que de rendre effectif l'engagement de notre pays à garantir aux femmes ce droit fondamental de choisir le moment de leur maternité, puisque, chacun ici en conviendra, il n'est pas concevable de défendre un droit sans s'attacher à lever tout ce qui peut faire obstacle à son libre exercice. Force est de constater que j'avais sous-estimé l'effet du calendrier électoral. La campagne présidentielle offre manifestement une formidable caisse de résonance à celles et ceux qui contestent le principe même du droit à l'IVG. Nous savions que les adversaires de la régulation des naissances n'avaient jamais vraiment désarmé, mais leur hostilité s'exprime de plus en plus ouvertement. Je le regrette, comme je récuse toutes les tentatives d'instrumentalisation de cette proposition de loi par celles et ceux qui entendent profiter de ce moment particulier pour reprendre leur combat contre l'IVG. Je veux donc rappeler brièvement l'unique objet du débat qui nous réunit cet après-midi : assurer, d'une part, la protection des usagers, en l'espèce des usagères, d'internet, d'autre part, l'accès au droit. Les enjeux sont clairs : garantir la fiabilité et la qualité des informations diffusées sur internet. Vous le savez, la Toile est aujourd'hui la première source d'informations relatives aux questions de santé pour les jeunes et les hommes, dans son rapport relatif à l'accès à l'IVG paru en 2013, rappelait ces chiffres issus du baromètre santé 2010 : dans cette tranche d'âge, 40 % des hommes et 57 % des femmes utilisent internet pour s'informer sur leur santé. Un tiers d'entre eux reconnaît que la consultation des sites spécialisés a modifié leur manière de se soigner et 80 % des plus jeunes estiment crédibles les renseignements qu'ils y recueillent. Internet constitue donc la première source d'information et d'orientation pour les femmes confrontées à une grossesse non désirée. Dès lors, il n'est pas acceptable, pas tolérable que des groupuscules anti-IVG y mènent impunément une nouvelle forme de propagande, sans dire clairement qui ils sont et ce qu'ils font.

dissimulés derrière des plateformes d'apparence neutre et objective qui imitent et concurrencent les sites institutionnels d'information, sites qui constituent souvent le premier recours des femmes qui souhaitent interrompre une grossesse.

Pis, elles sont parfois relayées par des cellules d'écoute animées par des militants sans aucune formation, qui prétendent aider et accompagner les femmes, alors qu'ils n'ont en réalité qu'un objectif : culpabiliser

et la véritable intention qui anime les « écoutants-militants » des numéros verts relayés sur ces plateformes. Chacun est évidemment libre d'exprimer son hostilité à l'avortement, je tiens à le redire, mais la diffusion de données orientées ou erronées production de témoignages négatifs et angoissants ne relèvent pas de la liberté d'information : il y a là, évidemment, une réelle volonté de tromper les femmes qui les consultent, une réelle volonté d'induire les femmes en erreur, de les faire douter et revenir sur leur décision. Je l'ai dit et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra : la liberté d'expression ne peut se confondre avec la manipulation des esprits. C'est cette duplicité qui constitue clairement une entrave au droit des femmes à disposer de leur corps. C'est donc à cette supercherie que nous avons aujourd'hui la responsabilité de nous attaquer. Depuis 2012, le Gouvernement lutte, avec constance et détermination, contre tout ce qui altère le droit à l'avortement. Garantir l'égal accès de toutes les femmes à l'IVG, quels que soient leur situation, leur âge ou leur lieu de résidence, est la priorité absolue qui nous a guidés. Avec le soutien de la majorité parlementaire, le Gouvernement s'est donc attaché à faciliter les démarches des femmes et à simplifier le parcours IVG, qui est aujourd'hui pris en charge à 100 %. Nous avons aussi renforcé l'offre de proximité, en donnant aux sages-femmes la possibilité de pratiquer des IVG médicamenteuses

Parallèlement, nous nous sommes attachés à améliorer l'accès des femmes à cette information essentielle avec de nouveaux outils, conformément aux recommandations formulées par le HCE le HCE : la création du site internet officiel ivg.gouv.fr ; l'ouverture, en septembre 2015, d'un numéro national d'information, anonyme, gratuit et accessible six jours sur l'année dernière de la première grande campagne gouvernementale d'information sur l'avortement, « IVG, mon corps, mon choix, mon droit ». Ces mesures ont incontestablement contribué à sécuriser l'exercice du droit des femmes à disposer de leur corps. Pour autant, vous le savez parfaitement, ces dispositifs ne parviennent pas à contrer efficacement l'offensive que les anti-choix mènent sur la Toile. À la faveur des usages croissants du numérique, et parce qu'ils se dissimulent sous l'apparence de la neutralité, ces sites touchent des

Les outils juridiques conçus pour combattre cette désinformation doivent donc être spécifiquement adaptés aux évolutions de la communication sur internet et sur les réseaux sociaux. C'est l'unique objectif de cette proposition de loi établir une nouvelle forme de délit d'entrave à l'ère numérique, pour compléter l'arsenal législatif qui sanctionne les actes visant à limiter l'accès à l'avortement et aux informations qui s'y rapportent. Que les anti-choix se rassurent : si cette proposition de loi est adoptée, ils pourront continuer en toute légalité à combattre l'IVG. Je tiens à le redire une fois encore : ces activistes ont parfaitement le droit d'être hostiles à l'avortement, de le dire, de l'écrire, de le revendiquer sur internet, dans la rue ou ailleurs. Cela relève de la liberté d'opinion et d'expression, qu'il n'est pas question de restreindre, contrairement à ce que certains essaient de faire accroire. C'est bien la désinformation, le mensonge et la manipulation des esprits organisés sur les plateformes et les lignes d'écoute que ce texte vise à sanctionner. les sénateurs, que vous partagiez cette exigence, et que vous soyez, toutes et tous, convaincus que le progrès technologique ne doit pas servir à mettre en danger ou à faire reculer les droits des femmes.

la nécessité de garantir l'accès des femmes à une information de qualité, à une contraception adaptée et à l'avortement sûr et légal » ; « l'importance du droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes en France, en Europe et dans le monde ». En conclusion, je veux vous alerter

Ce serait non pas une victoire des amis de la liberté, mais un point marqué par les anti-IVG. Pensez-y, mesdames, messieurs les sénateurs, au moment où vous nous menacerez d'une censure du Conseil

le Sénat avait adopté le 7 décembre dernier une rédaction remaniée de la proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. À la suite de notre vote, la commission mixte paritaire s'est réunie le 24 janvier. Elle n'a pu aboutir, ce que je regrette.

Il s'agit d'apporter une réponse à un problème grave et précis, celui que rencontrent nos concitoyens, parmi eux nos enfants, nos proches, face aux nouveaux moyens par lesquels s'exerce l'entrave à l'IVG, c'est-à-dire le numérique et les nouvelles technologies.

La navette parlementaire a repris son cours et les députés ont de nouveau examiné la proposition de loi, en commission le 25 janvier puis en séance le lendemain. Je relève d'emblée que le texte de l'Assemblée nationale a pris en compte plusieurs apports du Sénat. Il permet en effet désormais de viser l'ensemble des personnes cherchant à se renseigner sur l'accès pratique à l'IVG,

Les députés ont par ailleurs procédé aux coordinations que nous avions envisagées pour l'application du texte outre-mer. Cependant, le texte issu de l'Assemblée nationale vise explicitement l'entrave « par voie électronique ou en ligne et rétablit des éléments de caractérisation du délit que nous avions jugés plutôt inopportuns. Le texte adopté par le Sénat en première lecture avait permis de résoudre ces difficultés tout en préservant l'équilibre du droit actuel. Il permettait en effet d'atteindre l'objectif de la proposition de loi en changeant le droit en vigueur. La rédaction proposée par la commission des affaires sociales, je le rappelle, avait été adoptée par notre assemblée à une large majorité des suffrages exprimés. À l'issue de débats salués par l'ensemble des parlementaires pour leur qualité juridique et la possibilité donnée à chacun d'exprimer ses convictions, la proposition de loi que vous défendez, madame la ministre, avait ainsi été approuvée au Sénat par 173 voix, contre 126, sur les 299 votes C'est pourquoi j'ai proposé à la commission des affaires sociales, lors de notre réunion du 8 février dernier, d'adopter à nouveau le texte du Sénat voté en première lecture, en commission et en séance publique, position qui me semblait relever d'une grande cohérence. Curieusement, cette proposition de rétablissement n'a pas recueilli une majorité de suffrages. Une diversité de points de vue s'est exprimée. Certains ont estimé que ni le texte de l'Assemblée nationale ni celui du Sénat ne donnaient pleinement satisfaction. D'autres ont considéré que le Sénat était allé aussi loin que possible dans la recherche d'un compromis et que l'échec de la commission mixte paritaire devait marquer la fin de nos débats. Pour d'autres encore, le sujet est trop important pour que nous refusions d'en débattre. À l'issue de nos travaux, la commission des affaires sociales n'a adopté ni l'amendement de retour au texte du Sénat, que j'avais proposé par souci de cohérence, ni le texte de l'Assemblée nationale. En application de l'article 42 de notre règlement, nos débats portent donc sur ce dernier texte. Je respecte bien évidemment tous les points de vue qui ont été exprimés lors de notre commission, dont j'espère restituer fidèlement les travaux. Il me semble néanmoins que le Sénat avait apporté en première lecture une réponse proportionnée à une véritable question de société, l'enjeu étant de garantir l'effectivité d'un droit qu'aucun parmi nous ne conteste, celui de recourir à une interruption volontaire de grossesse. En raison d'un calendrier contraint, la première phase d'examen de cette proposition de loi a été particulièrement rapide. Elle a donc d'abord connu successivement plusieurs modifications importantes en peu de temps. peu de temps. Trois mois se sont écoulés depuis le début de nos travaux, et nous pouvons aujourd'hui considérer que nous avons mené, en commission comme en séance, un examen approfondi de ce texte. En tout état de cause, comme nous en étions convenus lors de nos débats en première lecture, le dispositif dont nous discutons n'a de sens que dans le cadre d'une politique de santé plus globale permettant l'égal accès de toutes les femmes à l'IVG et de toute personne à l'information sur celle-ci.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

à prendre des décisions qui peuvent être particulièrement graves et douloureuses pour elles. Recourir à l'IVG n'est jamais une solution de facilité.

la nouvelle lecture au Sénat de la proposition de loi sur le délit d'entrave numérique à l'IVG fait suite à l'échec de la commission paritaire, échec qui a mis en évidence toute l'ambiguïté de ce texte. texte. Le rapporteur, Stéphanie Riocreux, en a bien senti la légèreté juridique en proposant d'amender le texte de l'Assemblée nationale. Dans son rapport devant la commission des affaires sociales, le 8 février dernier, notre collègue légitime son amendement « par les par les éléments de caractérisation du délit juridiquement plutôt inopportuns, voire contre-productifs du texte de l'Assemblée Madame la ministre, en septembre dernier, vous avez qualifié d'artifice de procédure le non-examen, par la majorité sénatoriale, d'un amendement hors sujet

Votre indignation, madame la ministre, s'est égarée sur une prétendue ambiguïté sénatoriale, tellement peu avérée que je propose un amendement sanctionnant civilement les excès d'expression incompatibles avec la loi sur l'IVG, loi portée avec courage et humanité Mais votée grâce à la gauche ! ... qu'aucun sénateur centriste ne voudrait ou ne tenterait de remettre en cause. Madame la ministre, notre indignation à nous, sénateurs centristes, est suscitée par votre silence abyssal, sauf cet après-midi, sur l'insuffisance des actions de prévention. Si l'IVG est un droit, nul ne peut décemment oser affirmer qu'il s'agit d'un droit banal ou anodin. L'IVG ne saurait être considérée comme un moyen de contraception. À cet égard, l'insuffisance de la prévention relève d'une insouciance coupable, car elle touche les plus faibles, les plus fragiles dont la détresse avait inspiré Simone Veil. En effet, alors que dès 2013 le Haut Conseil à l'égalité avait émis dans un rapport un certain nombre de préconisations, pourquoi avoir attendu 2015 pour créer un numéro vert ? Pourquoi le site officiel du ministère de la santé est-il moins efficace que d'autres sites ? Pourquoi allouer des moyens insuffisants au planning familial, qui joue un rôle pourtant essentiel d'information sur la sexualité, la prévention, la contraception

qui, cumulée avec l'indignation du Gouvernement sur les amendements sénatoriaux traitant des abus d'expression numériques dans le cadre de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, apparaît quelque peu surréaliste et crée des doutes sur vos véritables intentions. La commission des lois, par la voix de notre éminent collègue Michel Mercier, a exprimé des doutes sérieux sur la compatibilité juridique du texte qui nous est proposé avec le droit français et européen, Elle est en contradiction avec la directive européenne du 8 juin 2000 sur les services de la société de l'information, qui encadre très étroitement les responsabilités pénales et la procédure d'interdiction au sujet des infractions en ligne.

et les moyens employés, qui constitue l'un des piliers de la jurisprudence de la Cour de justice. Permettez-moi de m'interroger : s'agirait-il, par ce texte, de donner un signe, un gage politique ? Dans ce cas, votre sanction est un leurre, qui se heurte au droit et aux principes constitutionnels qui fondent notre démocratie. Vous empruntez une voie dangereuse ; vous franchissez sans prudence le Rubicon de la liberté d'expression. Si vous être vraiment soucieuse d'efficacité et du respect des libertés démocratiques, vous ne pouvez pas choisir d'envoyer quelqu'un en prison pour des propos, aussi faux soient-ils, tenus sur un site librement consultable. Vous préférerez une écoute attentive de la proposition constructive de délit civil que je présenterai. Madame la ministre, le sujet dont nous parlons ne peut être l'otage d'un contexte électoraliste. Mme la

Dire est utile, mais, laisser croire qu'en nommant un problème on l'a résolu, c'est une faute. Le législateur n'est pas un porte-étendard au service d'une communication idéologique. Le législateur écrit la loi et garantit son applicabilité. Alors, fuyons définitivement toute ambivalence et toute ambiguïté, car si dire est utile, pouvoir faire vraiment est essentiel à la crédibilité politique. Pensez-y aussi, madame la ministre

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour combattre une nouvelle forme d'entrave à l'IVG. L'entrave a évolué et prend aujourd'hui la forme de sites internet extrêmement malveillants. Ces derniers

Il n'est pas possible d'accepter la diffusion d'informations mensongères sur le déroulement d'une IVG, sur les conséquences d'une IVG pour instiller le doute dans l'esprit des femmes à un moment où elles sont particulièrement vulnérables et se posent des questions. Déjà, en novembre 2013, un rapport du Haut Conseil à l'égalité observait « depuis quelques années une montée en puissance très importante de sites cherchant à tromper délibérément les internautes en se faisant passer, au premier abord, pour des sites purement informatifs ». Ces sites internet apparaissent bien souvent en tête des résultats des moteurs de recherche, surtout sur le plus usité, et parfois bien avant les sites officiels. Ils utilisent les mêmes codes couleur ou des éléments de langage similaires pour donner l'illusion de la fiabilité de leurs informations. Certains diffusent même des adresses erronées de centres du planning familial, ralentissant ainsi l'accès à ces établissements. Selon nous, toute atteinte au droit des femmes à disposer de leurs corps appelle une réponse à la hauteur des enjeux, qui doit donc se placer aussi sur le plan pénal.

ou même à l'action des pouvoirs publics en la matière, doit être sanctionnée. Face aux évolutions numériques, nous pensons donc, même si nous nous sommes posé des questions au début, qu'il convient de compléter l'arsenal législatif. Il faut le transposer du monde réel au monde numérique pour tenir compte de ce que les progrès techniques permettent de faire. La commission des affaires sociales du Sénat n'a pas adopté le texte sur lequel elle avait pourtant trouvé un consensus il y a quelques semaines. Il faudra nous expliquer ce qui, hormis de prochaines élections, justifie cette évolution.

La version du présent texte issue de l'Assemblée nationale rend applicable l'entrave numérique à l'IVG aux deux alinéas de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique. Elle concerne aussi bien l'entrave à l'accès aux établissements que l'entrave par le biais de pressions morales ou psychologiques. Cette rédaction, qui précise que l'entrave numérique concerne les indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif, nous paraît à la fois claire et posée. Elle est la mieux à même de répondre aux interrogations légitimes quant aux risques d'une atteinte à la liberté d'expression. l'avortement est un droit fondamental, et il est de notre devoir d'en garantir l'exercice par tout moyen ans après la loi Neuwirth, dont nous avons célébré l'importance il y a quelques jours, au Sénat, en présence de sénateurs et de sénatrices de tous les horizons, nous pensons que l'amendement qui vient d'être voté en commission tend à amoindrir considérablement le présent texte, et donc à lui ôter une partie de son sens.

dans des délais extrêmement contraints, sur un sujet aussi important, sans qu'un débat approfondi ait pu être tenu. C'est un scandale ! J'ai entendu ici ou là qu'il y avait, de notre part,

notamment non législatives, pouvaient permettre d'améliorer plus efficacement la diffusion de l'information sur l'IVG, étant précisé que nous souscrivons au constat sur la nécessité de cette information. le Gouvernement pourrait agir afin d'améliorer le référencement des sites officiels d'information au sein des moteurs de recherche sur internet. accélérée n'a pas permis d'avoir un avis du Conseil d'État sur des dispositions qui sont susceptibles de porter une atteinte substantielle à la liberté d'expression. Ces précisions Je l'ai déjà affirmé à cette tribune, mes convictions et ma pratique médicale me conduisent à défendre tout ce que les progrès de la science apportent à la liberté individuelle : je dis bien tout. Défendre une liberté, promouvoir un droit sans pour autant porter atteinte de façon insidieuse à un autre droit ou à une autre liberté, tel est le point d'équilibre que nous devons trouver en tant que législateur, équilibre essentiel au bon fonctionnement de nos sociétés démocratiques, à la fois si fragile- on le voit en ce moment -et si indispensable. Ce point d'équilibre repose sur le besoin de se sentir respecté dans ses convictions et dans l'exercice de sa liberté, et c'est sur lui que reposent notre contrat social et notre cohésion. cohésion. Madame la ministre, c'est bien là que réside toute la difficulté de ce texte. En effet, j'ai le sentiment que vous faites l'amalgame entre le fait d'empêcher

rapporteur pour avis, dans l'état actuel du droit, le délit d'entrave se caractérise par le fait qu'il doit être localisé à l'intérieur des établissements pratiquant l'IVG. deux hypothèses sont retenues. La première survient lorsque les personnels, médicaux ou non, ou les femmes qui souhaitent recourir à une IVG sont empêchés d'entrer ou de circuler dans ces établissements. La seconde est issue de l'élargissement du délit d'entrave assuré la loi de 2001 : elle concerne les pressions psychologiques exercées sur les femmes qui souhaitent subir une IVG ou sur leur entourage, mais toujours dans le cadre d'un établissement pratiquant l'IVG. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation admet assez facilement le délit d'entrave, mais toujours dans un cadre légal. Elle est fidèle en cela au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Or les dispositions de ce texte ne visent plus les agissements physiques qui se produisaient autour des centres d'IVG et pour lesquels le délit d'entrave a été instauré. Elles concernent certaines allégations diffusées sur internet ou directement auprès de personnes qui, après avoir consulté ces sites, prennent contact avec ceux qui les animent. Dans quelle mesure est-il envisageable de sanctionner pénalement des comportements qui prennent une forme tout à fait différente de ceux pour lesquels le délit d'entrave a été instauré ? Dans quels cas une telle situation devrait-elle justifier une réponse pénale ? Dans quelle mesure le délit d'entrave à l'IVG pourrait-il lui être transposé ? Et comment l'incrimination pourrait-elle être précisément définie ? Très objectivement, les réponses à ces questions ne paraissent pas évidentes. Pis, le texte adopté par nos collègues députés s'oppose à plusieurs principes, notamment constitutionnels. Michel Mercier l'a clairement démontré dans son rapport. Avec son autorisation, je me permets Avec son autorisation, je me permets de reprendre sa présentation. Pour ce qui est des principes généraux du droit pénal, ce texte contrevient, d'une part, au principe de clarté de la loi pénale et à l'objectif d'intelligibilité de la loi- en effet, ce texte est incompréhensible et Mme Riocreux, rapporteur de la commission des affaires sociales, l'avait elle-même qualifié, en première lecture, d'« inintelligible d'autre part, au principe de légalité des incriminations. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point est claire : le législateur doit aller au bout de sa compétence et définir pleinement les infractions, sans laisser au juge la liberté de le faire.

indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse » ne caractérise pas suffisamment une infraction.

d'une part, la liberté de recourir ou non à l'IVG, de l'autre, le respect de la liberté d'expression et d'opinion. Dans notre droit, la liberté d'opinion est clairement définie par le Conseil constitutionnel. Dans une décision du 11 octobre 1984, le juge constitutionnel estime que le législateur ordinaire ne peut porter atteinte à liberté d'opinion et d'expression que pour la rendre plus effective ou pour la rendre compatible avec une autre liberté de valeur constitutionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le droit de recourir à l'IVG est un droit, et non une liberté constitutionnelle. En effet, comment apporter la preuve irréfutable que la consultation des sites en question est l'élément déclencheur du renoncement au recours à l'IVG ? Au mieux, elle ne peut constituer qu'un élément supplémentaire dans une action en justice, mais je doute que cela aboutisse, ou nous entrerons alors dans une dimension inquiétante de restriction de la liberté d'expression Pourquoi avez-vous cette volonté de fragmenter, plutôt que d'aborder la question dans sa globalité en apportant des réponses différentes à des situations différentes, mais issues de la même origine : la numérisation de nos sociétés, la multiplicité des sources et la diversité des canaux d'information ? Ce texte, objectivement, ne résoudra rien ; il ne sert, une fois de plus, qu'à rouvrir les plaies. Madame la ministre, mes chers collègues, lors du vote de la loi Veil, le député Eugène Claudius-Petit, qui ne fit jamais mystère de ses convictions,

Nous le constatons bien, à trop vouloir répondre aux questions de société, par définition complexes et transversales, au moyen de mesures spécifiques et parcellaires, on ne résout rien, on ne régule rien, on ne pacifie rien. Or l'une des missions de la loi et du droit est précisément de réguler et de pacifier les relations sociales. Ce texte ne vise malheureusement pas cet objectif L'atteinte insidieuse que vous portez à cette liberté publique fondamentale ne risque-t-elle pas d'être le prélude à d'autres coups de boutoir ? Les bons sentiments ne suffisent pas à définir une politique. Notre rôle de législateur doit, bien au contraire, être synonyme d'efficacité et de prudence. Nous devons être toujours soucieux de préserver un équilibre entre la sauvegarde de la liberté d'expression et la nécessaire répression de ses abus. Pour l'ensemble de ces raisons, qui tiennent tant à la forme qu'au fond, au degré d'imprécision, source d'insécurité juridique à venir, à la précipitation, conduisant à un texte de circonstance non abouti, les élus du groupe Les Républicains voteront majoritairement contre cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire, nous examinons en nouvelle lecture la proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Pour parler de l'entrave opposée à un droit, il faut revenir sur le contexte dans lequel celui-ci s'exerce. Beaucoup d'évolutions ont eu lieu depuis la loi Veil, votée le 17 janvier 1975, reconnaissant le droit à l'avortement, à la suite d'une forte mobilisation des femmes et d'associations féministes et grâce à l'opiniâtreté d'une femme politique. Mais ce droit chèrement acquis a depuis été l'objet d'attaques de la part de conservateurs et d'intégristes religieux. Exercer un pouvoir sur le corps des femmes reste un enjeu fondamental. On constate une campagne sourde ou bruyante, selon le contexte politique plus ou moins favorable à l'émancipation humaine, mais constante et déterminée contre la loi Veil. Ainsi, à quelques mois de l'élection présidentielle, plusieurs conceptions s'affrontent, dont une vision nataliste de la société au nom d'un modèle unique de la famille,

convictions l'ont conduit à voter contre le remboursement de l'IVG par l'assurance maladie dès décembre 1982, contre l'allongement du délai à douze semaines de grossesse en juillet 2001 et contre la suppression du délai de réflexion en janvier 2016. C'est la vérité

le droit à l'interruption volontaire de grossesse a été remis en cause en Espagne en 2014 et plus récemment en Pologne. C'est une fois de plus les mobilisations nationales et internationales qui ont fait échouer ces projets funestes. En Italie, le pape François poursuit lui aussi son combat contre l'avortement en utilisant des mots d'une rare violence. Quant à la victoire de Donald Trump à la présidence de la première puissance mondiale, elle n'a rien pour rassurer Le nouveau président des États-Unis affirme vouloir « punir les femmes » pratiquant un avortement « illégal ». Il a signé un décret interdisant le financement d'organisations non gouvernementales internationales qui soutiendraient l'avortement. À cela s'ajoute la nomination à la Cour suprême du juge William Pryor, qui considère que « l'avortement est la pire abomination de l'histoire du droit. Deux millions de femmes se sont rassemblées, lors de « la marche des femmes » aux États-Unis, pour protester contre ces reculs. Dans toutes les capitales, des marches de solidarité ont eu lieu au lendemain de l'élection de Donald Trump. Face à cette remise en cause d'un des droits fondamentaux des femmes, il est indispensable de transformer le droit à l'avortement en un droit inaliénable. À travers la contre-offensive sur l'IVG se joue un bras de fer entre les partisans de l'émancipation humaine et ceux qui continuent à penser que les femmes sont d'éternelles mineures. Le combat des commandos anti-IVG a changé de terrain ; il se livre aujourd'hui sur internet et il est impératif d'apporter une réponse adaptée aux évolutions de notre société. Le délit spécifique d'entrave à l'IVG, créé en 1993, étendu aux violences morales depuis 2001 et notamment aux pressions morales et psychologiques, doit être étendu aux sites internet qui prétendent apporter une information neutre sur l'accès à l'IVG, alors qu'en fait ils font tout pour décourager les femmes de pratiquer un avortement. En réalité, on est face à une entreprise de désinformation qui instrumentalise le désarroi de femmes souvent jeunes et dans une situation Lorsque l'on sait qu'une femme sur trois a recours à une IVG au cours de sa vie, on mesure combien il est important d'informer et d'assurer l'accompagnement de ce choix. Contrairement à ce que certains laissent entendre, aucune femme ne prend la décision d'avorter le coeur léger. Assurer l'information et l'accompagnement des femmes ayant recours à une IVG, cela signifie effectivement lutter contre la manipulation des esprits par des sites de désinformation. Et que l'on ne prenne pas le prétexte de la liberté d'information ! Il me semble que le Sénat avait bien travaillé en première lecture

puisse exercer ce droit partout sur le territoire. Il faut conforter et renforcer les mesures que vous avez prises avec Mme Touraine. Je rappelle qu'en dix ans 130 centres IVG ont fermé, tandis que le nombre d'avortements est resté stable. Cela signifie que des femmes sont obligées d'aller avorter à l'étranger pour avoir une place dans les délais légaux. Selon Mme Véronique Séhier, coprésidente du planning familial,

il est impératif de maintenir les subventions aux associations qui militent au quotidien auprès des femmes et qui subissent des politiques de restrictions autant que des coupes franches. Je pense par exemple à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a réduit de 30 % la subvention accordée au planning familial.

On le voit, pour défendre le droit à l'avortement, il est nécessaire de créer les conditions pour que chaque femme ait accès aux mêmes informations, aux mêmes structures, aux personnels de santé compétents et bien formés. En conséquence, il faut déjouer les manoeuvres de sites peu peu scrupuleux qui, au nom de la liberté d'information, n'hésitent pas à désinformer pour faire prévaloir des convictions personnelles et empêcher les femmes de prendre leur décision en toute connaissance de cause. Pour toutes ces raisons, je déplore que nous n'ayons pas pu nous mettre d'accord en commission sur le vote consensuel auquel nous étions parvenus en première lecture.

effectif le plus rapidement possible dans l'intérêt des femmes. Mes chers collègues, je vous demande de réfléchir à ce que nous avons pu faire en première lecture et d'en tirer les conséquences pour voter majoritairement la proposition de loi qui

nous examinons en nouvelle lecture la proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire.

à l'information sur l'IVG en modifiant le délit d'entrave tel qu'il existe dans notre droit. Cet échec est regrettable, car nous avons toutes et tous la conviction que les femmes ont droit au respect de leur libre arbitre, hors de toute manipulation, de toute duplicité et de toute violence, pour décider d'interrompre ou non une grossesse avant la douzième semaine. personne ne remet en cause la nécessité du délit d'entrave tel que le législateur l'a défini en 1993, puis étendu aux formes de plus en plus sophistiquées de l'entrave à l'IVG. Nous partageons ces constats et ces convictions. Pourtant, nous ne sommes parvenus à un accord ni avec l'Assemblée nationale ni au sein de notre commission. Il semble que l'obstacle au compromis soit notre appréciation divergente de la portée de la proposition de loi en matière de liberté d'expression. Ce point mérite quelques éclaircissements. Toutes et tous, dans cet hémicycle, avons la conviction que la liberté d'expression est fondamentale, parce qu'elle est la condition d'exercice des autres libertés. Avec la liberté de conscience, la liberté d'expression est le socle de notre société pluraliste et tolérante, donc de notre démocratie. Fidèles à la philosophie de Voltaire, nous pouvons dire Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » Mes chers collègues, le texte qui nous est proposé ne remet pas cela en cause. En effet, les problèmes auxquels sont confrontées les femmes qui apportent leur témoignage sur les entraves à l'IVG ne sont pas les propos publics des mouvements anti-IVG,

sont les manifestations de la liberté d'expression et de conscience ; légitimement protégées par le droit constitutionnel et par le droit européen, elles ne sont en rien concernées par la présente proposition de loi. les problèmes, ce sont l'intimidation, la duperie, la violence psychologique, parfois le harcèlement qui s'exerce notamment au travers des mises en relation téléphonique des sites d'information. À ce stade- les témoignages recueillis sont éloquents la diffusion d'une information ou de l'expression d'une opinion, mais bien de la volonté de contraindre psychologiquement ses interlocuteurs. Pour les militants qui se cachent derrière ces sites et plateformes d'appels, il n'y a pas de Voltaire qui tienne Bien au contraire, leur approche est claire : « Je ne suis pas d'accord avec vous qui pensez à avorter, aussi, je vais me battre jusqu'au bout pour vous empêcher d'être en situation d'agir, car mes convictions doivent triompher de vous. Empêcher ces personnes de nuire est une nécessité et n'a rien à voir avec la liberté d'expression, qui n'a jamais inclus le droit d'imposer ses idées à autrui, encore moins par la contrainte ou la violence. Les tribunaux ont rappelé à plusieurs reprises qu'il ne saurait être question de liberté d'expression ni de liberté de conscience lorsque des militants anti-IVG bloquent les accès aux établissements, intimident le personnel médical ou font irruption dans la salle d'attente du planning familial pour imposer leurs prières. Dans une affaire jugée en 2015 par la Cour de cassation, un homme, après s'être introduit dans un centre du planning familial, a remis par surprise des chaussons de bébé à une femme venue recevoir des conseils pour une éventuelle IVG. Liberté d'expression ? Liberté de conscience ? Non, répondent la cour d'appel et la Cour de cassation : il s'agit là de pressions psychologiques et même de violences morales. Aujourd'hui, ces pressions, violences et menaces ne s'exercent plus seulement dans les établissements de santé ou au sein des centres du planning familial. Aujourd'hui, ces techniques d'entrave ont migré vers internet et les plateformes téléphoniques. Notre droit doit s'adapter à cette nouvelle modalité du délit d'entrave. C'est pourquoi cette proposition de loi prévoit que l'entrave à l'IVG doit être poursuivie y compris lorsqu'elle est commise à distance, par téléphone, internet ou textos, à la condition que soient réunis les éléments de sa définition, qui, eux, n'ont pas changé. Il faut rappeler que les éléments constitutifs du délit d'entrave ne sont pas remis en cause : tel qu'il est proposé par l'Assemblée nationale, le nouveau chapeau de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique implique que la « diffusion ou transmission d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences d'une IVG sera constitutif de délit d'entrave si et seulement si cette diffusion a conduit à la perturbation de l'accès à un établissement ou si elle a atteint l'intensité d'une menace, pression morale ou intimidation. Ce point est important et suscite beaucoup d'incompréhension, car la rédaction issue de l'Assemblée a fait craindre à certains que le chapeau de cet article ne puisse être mis en application par les juges indépendamment du 1° et du 2° de son texte. C'est pourquoi, dans un souci de compromis, le groupe socialiste

Nous y sommes presque ! Mme la rapporteur a apporté sa précieuse contribution, et c'est dans cet esprit de compromis, autour de fortes convictions partagées en faveur de l'émancipation des femmes, que le groupe socialiste et républicain votera la nécessaire modernisation du délit d'entrave.

dans un contexte international de montée de l'obscurantisme et des extrémismes religieux qui menacent les droits fondamentaux des femmes, notamment leur liberté de disposer de leur corps et de maîtriser leur fécondité. Je vous avoue, mes chers collègues, que j'éprouve un sentiment d'inquiétude et de révolte devant les attaques répétées contre les droits des femmes dans de très nombreux pays,

le gouvernement polonais a tenté d'interdire à nouveau l'avortement. La première décision prise par le président Trump a été un décret interdisant le financement d'organisations non gouvernementales internationales soutenant l'avortement. Il y a quelques jours,

Quelle tradition, mes chers collègues ! C'est vrai ! Souvenons-nous qu'en 2013 le gouvernement espagnol avait approuvé un avant-projet de loi interdisant l'avortement, avant de renoncer sous la pression de dizaines de milliers de manifestants descendus dans les rues. rues. Si ce retour des attaques à l'encontre des libertés des femmes ne peut que susciter notre inquiétude, il met en lumière,, l'action forte d'hommes et de femmes qui se battent pour préserver des droits durement acquis acquis au cours de l'histoire. Ainsi, la marche noire des militantes polonaises de l'association Sauvons les femmes a contraint leur gouvernement pour le moment, à ses velléités conservatrices, ce qui leur a valu de recevoir le prix Simone de Beauvoir. Nous sommes quelques-unes dans cet hémicycle à avoir contribué à les faire venir à Paris, le mois dernier, pour recevoir ce prix, tant leur mobilisation a suscité notre admiration et nous appelle à mener, ici, dans le pays des droits de l'homme, une véritable bataille

en utilisant des arguments nauséabonds. Ainsi, les femmes se serviraient-elles de l'avortement comme d'un moyen de contraception, sans aucun état d'âme ! mes chers collègues, que cet acte, avec tout ce qu'il implique dans la vie d'une femme, puisse être abordé avec une telle légèreté par celles qui en font le choix ? Le traumatisme, aussi bien physique que psychologique, est une réalité ; prétendre l'inverse serait un dangereux mensonge. Nous devons lutter contre la diffusion de telles idées,

portée aux droits des femmes constitue un recul pour la société tout entière, chacune des idées conservatrices traversant le débat public

été comprise. Nous proposons effectivement de sanctionner des propos absolument incompatibles avec la loi sur l'IVG, mais l'on ne saurait mettre en prison des gens pour une expression sur des sites librement consultables ni confondre des violences physiques à l'encontre des femmes qui cherchent à se renseigner et des propos, aussi faux soient-ils, tenus sur internet. Enfin, il convient de respecter le principe de proportionnalité. Madame la ministre, j'ai été

Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, sur lequel nous nous étions tous accordés. La rédaction proposée permet de rétablir la distinction nécessaire entre l'objectif poursuivi par les auteurs du délit, qui figure dans le chapeau actuel, et les moyens par lesquels il est constitué, à savoir l'entrave physique, d'une part, et l'entrave psychologique ou morale, d'autre part. Cette rédaction implique sans ambiguïté que la communication électronique fait partie des moyens par lesquels peuvent s'exercer les pressions et les menaces constitutives constitutives du délit d'entrave. Enfin, par rapport au texte actuel, elle précise que les personnes cherchant à s'informer sur l'IVG, notamment sur internet, peuvent être reconnues victimes de ces pressions. Le texte actuel du code de la santé publique ne vise que les personnes se trouvant dans les établissements de santé ou dans les centres pratiquant des IVG. Cet amendement tend, par ailleurs, à procéder aux coordinations nécessaires à son application en outre-mer.

que rapporteur, je ne suis pas totalement certaine que nos débats aient été tout à fait clairs. Je me permets donc de rappeler les raisons qui avaient conduit au rejet en première lecture. La proposition de loi ne crée pas un délit nouveau, mais s'inscrit dans le cadre du délit d'entrave par voie psychologique, lequel existe depuis 2001.

par notre droit. Pour plusieurs raisons, nous nous opposons à son adoption. Tout d'abord, il est totalement inopportun de complexifier le droit en matière d'information et d'accès à l'IVG en juxtaposant dans le code de la santé publique une sanction civile et une sanction pénale. Soit il y a entrave, c'est-à-dire volonté de priver quelqu'un de son droit,

désinformer, mentir, tromper pour imposer une grossesse à une femme qui n'en veut pas parce que ça n'est pas son projet de vie, c'est aussi lui infliger une violence.

mais ce n'est pas parce que l'on est contre l'IVG que l'on a le droit de tromper, de mentir, de désinformer, d'exercer des pressions sous couvert d'une information faussement neutre, dans l'objectif de dissuader les femmes d'y recourir.

que de l'aide et des conseils. Nous voulons simplement lutter contre les effets de la tromperie, de la manipulation, de la désinformation et protéger le droit des femmes de s'informer objectivement. Nous entendons protéger leur liberté

l'autre, du groupe de l'UDI-UC. Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

majoritairement l'amendement qui nous est présenté par Patricia Schillinger.

explication de vote. Chaque liberté gagnée mérite d'être défendue, non seulement pour nos compatriotes, mais aussi en souvenir de ceux qui ont lutté pour les obtenir.

encore une fois qu'un compromis utile n'ait pu être trouvé afin que le Sénat et l'Assemblée nationale apportent une réponse commune aux inacceptables manifestations contemporaines du délit d'entrave à l'IVG. Les femmes attendent du législateur une réponse ferme, une réponse susceptible de les protéger de ceux qui portent atteinte à leur libre arbitre et, en définitive, n'acceptent pas qu'elles aient le droit de disposer de leur corps. C'est le moins que l'on puisse faire, cinquante ans après l'adoption de loi Neuwirth, qui a donné aux femmes le droit à la contraception, ouvrant une ère nouvelle de la grande histoire des femmes, une ère où les grossesses non désirées ne seraient plus leur lot commun, leur fatalité. Ce fut en effet un moment historique. La sociologue Françoise Héritier rappelait en 2002, dans son ouvrage qu'une enquête qu'une enquête d'opinion avait à l'époque interrogé les hommes et les femmes pour savoir quels étaient à leurs yeux les principaux événements du XX siècle. Les femmes avaient placé en premier, à 90 %, le droit à la contraception, les hommes, majoritairement, la conquête de l'espace ... Peut-être venons-nous vraiment de planètes différentes ! Mais aujourd'hui, ensemble, nous devons conforter le droit des femmes et répondre aux entraves dont elles sont la cible. Je remercie vivement M. Roche et tous

La séance est reprise.

Monsieur le sénateur, une telle manifestation d'amitié et d'empressement justifie que je fasse un effort pour vous être agréable. Aussi, il est normal que, sur la question de la présence des services publics en milieu rural, question importante Nous sommes tous, quelles que soient nos appartenances et nos sensibilités politiques, dans l'obligation de redresser nos comptes. Nous ne les redresserons pas si nous ne faisons pas un effort de maîtrise des effectifs de la fonction publique locale et territoriale. Je le sais, nous sommes dans une période électorale,

Les efforts budgétaires réalisés, qui ont permis de diminuer le déficit de l'État- nous atteindrons nos objectifs de déficit public cette année -, ne nous ont pas empêchés de créer des postes là où des priorités Vous avez évoqué la suppression de postes dans la police et la gendarmerie. Je veux rappeler- vous auriez pu le dire dans votre question, car je sais votre grande rigueur intellectuelle -que nous avons créé 9 000 postes

Le deuxième point sur lequel je veux insister- vous le savez parfaitement puisque je me suis rendu dans votre département, accompagné des élus, dont vous-même -concerne les préfectures et sous-préfectures

en mettant en place le plan Préfectures nouvelle génération, qui conduit à faire des efforts par la création de plateformes de titres. Cela permet de réinjecter dans les préfectures et sous-préfectures des effectifs nouveaux. Les effectifs

et une relocalisation de la gendarmerie, qui profite d'ailleurs de cette relocalisation pour bénéficier de la modernisation de locaux, nous sommes dans le confortement du maillage territorial. Monsieur le sénateur, je vois dans votre question l'expression, au travers de la faconde et de la fougue qui vous caractérisent, d'une volonté de précision que je vous apporte bien volontiers. Vous pourrez ainsi rentrer dans votre département rasséréné et rassuré, j'en suis convaincu,

L'actualité du nucléaire est cette semaine particulièrement dense. L'incident de la semaine dernière à Flamanville, troisième incendie dans une centrale en dix jours- deux à Cattenom et un à Flamanville -, rappelle que le risque zéro n'existe pas et souligne tout particulièrement la fragilité de nos installations vieillissantes. Pendant ce temps, personne ne sait vraiment où sont passés les noyaux fondus de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, qui se sont fait la malle en perçant un trou dans la dalle de béton, mais qui se rappellent à notre bon souvenir par des radiations intenses. Le dernier rapport de TEPCO, l'exploitant de la centrale, annonce ainsi des taux de radiation dans le réacteur numéro 2 de nature à tuer immédiatement tout individu s'en approchant. La catastrophe est bel et bien aussi économique. À l'échelle mondiale, le conglomérat industriel japonais Toshiba, après une perte de plus de 3 milliards d'euros liée à sa filiale nucléaire Westinghouse, a annoncé ce mardi qu'il allait limiter les risques dans l'activité nucléaire à l'étranger, en ne prenant plus en charge la construction de nouveaux projets. Il se désengage même de l'Inde, que certains dépeignent pourtant en eldorado du nucléaire. En France, cet échec économique est aussi patent. La publication des résultats annuels d'EDF montre une baisse de près de 15 % de son résultat net courant, avec un négatif de 1,6 alors que ce qu'il est convenu d'appeler le mur d'investissement- Hinkley Point, grand carénage des centrales existantes, reprise d'Areva moribonde, et j'en passe -se rapproche, lui, à toute vitesse. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, impute une large part de ce résultat à la baisse des prix du marché, dans un contexte de surproduction et il a donc de nouveau demandé une hausse des tarifs de l'électricité. Madame la ministre, pour cette dernière question avant la fin de cette session, connaissant votre liberté de ton, pouvez-vous nous dire, en toute liberté puisque ce n'est vraisemblablement pas ce gouvernement qui sera chargé de cette décision, si vous considérez vous aussi, comme M. Lévy, inéluctable l'augmentation des prix de l'électricité en France pour faire face aux coûts d'investissement dans le nucléaire ou pensez-vous qu'une autre voie est possible ?

de l'électricité en France globalement et au niveau mondial. Grâce à cette réforme, depuis plus de dix ans, les tarifs adoptés au 1 août 2016 ont baissé en moyenne de 0,5 % pour les particuliers et de 1,5 % pour les artisans.

les raccordements d'éoliennes ont augmenté de 45 % au cours de l'année qui vient de s'écouler. Par conséquent, on peut dire que c'est grâce aux énergies renouvelables qu'il n'y a pas eu de coupure de courant pendant le pic de froid dans la mesure où neuf réacteurs nucléaires

Je me réjouis de voir qu'EDF devient un opérateur très important des énergies renouvelables et des énergies alternatives, puisqu'il investit 2 milliards d'euros dans cette filière

À l'heure où les enjeux sur l'approvisionnement et la transition énergétique sont des plus importants, comme on vient de l'entendre, à l'heure où la question de la sécurité nucléaire se pose avec acuité, au moment où des milliers de nos concitoyennes et concitoyens sont privés d'électricité à cause des tempêtes et où les agents EDF sont à pied d'oeuvre, c'est une véritable imposture à laquelle se prépare la direction d'EDF ! Alors qu'elle a entamé plusieurs chantiers industriels de grande ampleur et après déjà de nombreuses suppressions de postes au fil des années- l'an dernier -, ce ne sont pas moins de 5 000 nouvelles suppressions qui sont annoncées par le président de cette belle entreprise publique, soit 7 % de l'effectif ! Tous les secteurs seront touchés, la recherche et le développement ne sont pas épargnés et, dans mon département, les agents des boutiques EDF m'ont déjà alertée. EDF doit avoir les moyens d'assurer le service public de l'électricité dans la durée. Elle doit être le pivot de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables, alors que l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques la prive de la première d'entre elles. EDF, belle entreprise publique, à l'instar de l'ensemble de nos services publics, doit être présente sur tous nos territoires. Madame la secrétaire d'État, quand l'État aura-t-il une politique industrielle et énergétique de long terme cohérente et déconnectée des enjeux financiers ? Quand jouera-t-il son rôle de stratège pour assurer la sécurité des approvisionnements, notre indépendance énergétique et la préservation de nos savoir-faire irremplaçables ?

ce sont des mesures d'incitation au départ sur la base du volontariat. Il ne s'agit donc pas de licenciements ; je tiens à souligner ce point essentiel pour les salariés de l'entreprise. Deuxièmement, sont prévus des non-remplacements de départs en retraite, qui correspondent à environ 6 % des effectifs d'ici à 2019. Ces non-remplacements font également suite à des recrutements ayant eu lieu entre 2011 et 2016- ils ont été de l'ordre de 20 000 -, conduisant à un accroissement des effectifs

Dans ce contexte, le Gouvernement soutient l'effort réalisé par l'entreprise. En effet, le 22 avril dernier, le Gouvernement a indiqué qu'il soutenait le plan stratégique d'EDF dans la production d'électricité décarbonée, le programme CAP 2030, dans le cadre d'efforts partagés entre l'État et l'entreprise. Ainsi, un programme d'investissements particulièrement important a été décidé, financé notamment par une augmentation du capital de 4 milliards d'euros, dont 3 milliards apportés par l'État, qui accepte également de percevoir ses dividendes en actions pour deux années supplémentaires. EDF s'est, de son côté, engagée, dans le cadre de ce plan, à faire des efforts concernant ses charges, à maîtriser ses investissements et à céder des actifs.

Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs jours, à la suite de l' « affaire Théo », qui a suscité une émotion légitime, des violences urbaines ont éclaté en région parisienne. Ce phénomène n'est pas nouveau, malheureusement, puisque nous le connaissons depuis plus de dix ans. mes chers collègues, la répétition ne doit pas forcer l'acceptation : ces violences sont inacceptables, comme l'a redit le Président de la République ce matin. Au nom de mon groupe, je tiens ici à les condamner. L'ordre républicain doit être rétabli dans les banlieues,

et les citoyens. Rétablir cette confiance sera indispensable au moment où certains ont l'esprit qui s'embrase : ne rien céder aux casseurs, mais aussi ne rien céder à l'extrême droite, qui souffle sur les braises par ses déclarations de divisions. Dans ce contexte, les polémiques doivent être évitées, mes chers collègues. Seules la justice et la sécurité comptent ! La réponse de l'État doit être ferme, à la hauteur des mots du jeune Théo, qui avait appelé avec sang-froid et courage à l'apaisement la semaine dernière. Il a montré une grande responsabilité, dont quelques-uns devraient s'inspirer avant de créer des polémiques à des fins bassement électorales. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit ce matin, la reconstruction de la police est et sera longue. La reconstruction du lien entre les citoyens et ceux qui les protègent sera aussi longue, nous le constatons tous les jours. Mais il est une chose urgente : le rétablissement de la sécurité dans les banlieues, où les populations n'en peuvent plus. Mes questions sont donc les suivantes : quelle est l'action de l'État face aux événements actuels pour rétablir l'ordre dans toutes les banlieues ? Comment rétablir demain la confiance entre citoyens et police ?

il faut poser des principes simples, clairs et fermes. Ces principes, je veux les énoncer devant le Sénat cet après-midi. Premier principe : aucune violence, d'où qu'elle vienne, dans les quartiers et partout ailleurs sur le territoire national, ne saurait être tolérée. Aucune violence n'est jamais tolérée par ceux qui sont chargés de la direction des forces de police et de gendarmerie. Nous avons été maintes fois interpellés dans cet hémicycle et à l'Assemblée nationale sur les événements survenus sur l'autoroute A1 ou à Moirans. Chaque fois, nous avons eu droit au même discours : l'autorité de l'État ne serait pas respectée sous prétexte que des actes violents auraient été commis de la part d'individus qui n'hésitent pas à enfreindre la loi en convoquant la violence. Chaque fois, le Gouvernement a apporté la même réponse : le droit passera ; la justice passera ; les individus seront interpellés, ils seront jugés, et ils le seront sévèrement.

pour élucider, enquêter et procéder à l'interpellation de ceux qui enfreignent la loi. Quand on est républicain, attaché à l'autorité de l'État et au au principe de l'État de droit, on ne fait pas une polémique par jour ; on manifeste son attachement au droit et on rend hommage aux forces de sécurité qui, quotidiennement, sur le terrain, accomplissent la mission difficile qui est la leur avec courage et dévouement, comme doit remplir sa mission tout service public. Deuxième principe, sur lequel je veux insister : les relations entre la police et la population- c'est aussi cela l'État de droit -doivent être empreintes d'un respect mutuel. Nul ne peut accepter s'il est républicain, attaché à la fermeté et à l'État de droit, qu'il y ait quelque geste déplacé que ce soit qui soit condamnable et qui représente une forme de remise en cause des principes déontologiques auxquels la police doit se conformer. Lorsqu'il y a une remise en cause de ces principes, l'inspection générale de la police nationale est saisie en administratif et en judiciaire : elle permet aux juges de faire leurs enquêtes et de dire le

comme cela a été fait avec la remise en cause du Renseignement territorial. C'est ce gouvernement qui aura créé 9 000 postes dans la police et la gendarmerie, qui aura augmenté de 15 % les crédits accordés aux forces de sécurité, qui aura reconstitué le Renseignement territorial, ... Ça suffit les rémunérations des policiers et des gendarmes. L'autorité de l'État suppose aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, de donner des moyens à ceux qui oeuvrent en première ligne contre le terrorisme et l'insécurité, et pour l'État de droit. Enfin, le dernier point sur lequel je veux insister et qui me paraît, dans le contexte particulier où nous nous trouvons, le plus important : quand l'extrême droite est à ce niveau d'intentions de vote, ... La faute à qui ? ... la responsabilité que nous devons partager, ce n'est pas de souffler sur les braises en étant dans les responsabilités politiques, c'est de faire en sorte jour après jour que chaque parole prononcée

Monsieur le Premier ministre, il y a dix jours se déclenchait l'affaire Théo, du nom d'un jeune homme qui a été victime de violences policières. Disons-le d'emblée, la justice devra faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois,

Les scènes de violences urbaines des derniers jours inquiètent nos concitoyens à juste titre, car elles viennent s'ajouter à la menace terroriste, qui, de son côté, ne faiblit pas. La manifestation de dimanche dernier à Bobigny était annoncée, et elle était légitime. Mais les débordements qui ont suivi étaient, eux, inacceptables. Dans un contexte où le risque d'infiltration de casseurs violents, souvent très jeunes, est avéré, nous nous interrogeons sur le dispositif que vous avez mis en place. Pourquoi autoriser ce rassemblement si les risques de débordement étaient si importants ? Quels moyens étaient-ils mis en oeuvre pour en assurer le déroulement pacifique ? Comment se fait-il que ni le palais de justice de Bobigny ni les abords de la manifestation n'aient pu être mieux sécurisés ? Bref, quelle anticipation ? Les principes que vous avez énoncés, monsieur le Premier

aujourd'hui dans notre pays, singulièrement dans nos quartiers. Ceux-ci peuvent donner lieu à des manifestations. Je souhaite le dire ici de la façon la plus claire qui soit : il existe un droit à manifester dans notre pays quand cette manifestation est pacifique. En cas de manifestation, il doit y avoir protection, protection de la manifestation et des biens aux abords. En Seine-Saint-Denis, depuis le 4 février, ce sont 2 700 personnels qui ont été engagés dans le cadre du dispositif anti-violence.

Les forces de l'ordre ont été prises à partie, des véhicules incendiés, des bâtiments publics dégradés. Une patrouille a même dû se réfugier en toute hâte dans un commissariat. En effet, ce sont bien les policiers et tous ceux qui représentent l'État qui sont dans le collimateur des voyous.

Des milliards d'euros ont été déversés sans que rien ne change : on a tenté d'acheter la paix civile et l'État a renoncé à imposer son autorité. Votre seule réponse, nous la connaissons : il faut des moyens, toujours plus de moyens,

vous poserez-vous enfin les vraies questions, au lieu de vous contenter de pleurer sur les moyens perdus ou le manque de moyens à venir ?

Le monde est aujourd'hui rempli d'incertitudes. Quelle politique entend conduire le nouveau président des États-Unis ? Quelles sont les intentions du président Poutine ? Le terrorisme international influe, notamment, sur les politiques intérieures des pays occidentaux, soit en raison des menaces qu'il fait peser, soit en raison des déplacements de populations qu'il provoque. Et je ne parle pas de la Turquie, de la Corée du Nord ou de l'Iran, du réarmement de la Chine ou de la situation dans la bande sahélo-saharienne. On se dit que l'Europe devrait, pourrait être un pôle de stabilité, d'influence, mais on la sent quelque peu paralysée par ses peurs et le rejet qu'elle pourrait susciter en son sein. Le Brexit est là pour le rappeler.

du Benelux. Monsieur le Premier ministre, vous étiez à Berlin il y a quelques heures encore. J'aimerais que vous nous éclairiez sur les relations franco-allemandes, aussi nombreuses qu'étroites : le traité de l'Élysée et l'intelligence politique n'y sont pas étrangers. Cependant, on peut s'interroger sur la solidité de ce couple franco-allemand quand le contexte est au mieux chaotique, au pire hostile. Qu'en est-il des relations entre nos deux pays ? Qu'en est-il de leurs échanges ?

En matière de défense, les déclarations du président Trump sur la prise en charge par les Européens de leur propre défense conduisent-elles Allemands et Français à réfléchir à des initiatives communes, incitent-elles nos amis Allemands à s'engager davantage pour jeter les bases d'une Europe de la défense Monsieur le sénateur, je rentre effectivement à l'instant d'un déplacement à Berlin, où j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la Chancelière, le ministre des affaires étrangères et le président du Bundestag, ainsi qu'avec une délégation de parlementaires.

dans, cette magnifique phrase du commissaire européen Pierre Moscovici : « Économiquement, il faut se libérer de la menace de l'endettement

C'est sous ce gouvernement qu'ont été accomplis les efforts nécessaires au rétablissement des comptes publics

Le premier jour de ce même mois, le Gouvernement ouvrait un centre destiné à accueillir des « jeunes volontaires en phase précoce de radicalisation »- en clair, un centre aéré pour apprentis djihadistes

et républicain. Ma question s'adresse à Mme la ministre des outre-mer et concerne la situation de l'usine sucrière de Marie-Galante. Madame la ministre, à quelques jours du démarrage de la récolte, les planteurs de canne et la population de Marie-Galante vivent une situation très angoissante du fait des incertitudes pesant sur la prochaine campagne sucrière. L'État, qui s'est engagé à allouer une subvention de 1,6 million d'euros dans le cadre d'un projet industriel, subordonne le versement de cette somme à la continuation d'un accord passé avec un opérateur dont la technologie n'est plus en phase avec les objectifs environnementaux de la COP 21 et de la COP 22. Vous l'aurez compris, la culture de la canne et la production de sucre sont les poumons d'une économie alimentée par la seule unité sucrière en activité à Marie-Galante, le taux de chômage culmine à plus de 30 % et où la population est passée de 30 000 habitants en 1960 à moins de 12 000 en 2016. C'est dire combien l'avenir de l'île de Marie-Galante

Au nom des planteurs et de la population, dont je partage pleinement l'inquiétude et relaie les craintes, je vous demande solennellement, madame la ministre, d'organiser une rencontre avec l'ensemble des partenaires et, surtout, de procéder au déblocage de cette subvention, afin d'éviter une profonde crise économique et une tragique explosion sociale sur le territoire. La parole est à Mme la ministre des outre-mer. Monsieur

Compte tenu des contraintes spécifiques à l'île de Marie-Galante, la sucrerie doit faire face à des défis économiques et environnementaux particulièrement importants.

Toutefois, sa mise en oeuvre n'obère en rien le développement de l'initiative « Marie-Galante, l'île du tourisme durable » soutenue par la communauté de communes. Je suis convaincue que les deux projets ne sont pas concurrents mais compatibles, puisque la centrale thermique d'Albioma peut s'intégrer dans le projet plus global de la

1,6 million d'euros dès qu'un accord aura été trouvé sur le terrain. Une réunion s'est tenue lundi dernier entre le conseil départemental, le conseil régional et la préfecture : je souhaite qu'un consensus puisse se dégager dans les prochains jours. Madame la ministre, il faut lever les incertitudes qui pèsent sur l'ouverture de la campagne sucrière.

Il y a quelques mois, au nom du département de l'Aube, et plus particulièrement du Bar-sur-Aubois, j'ai fait observer qu'il y avait une contradiction formelle entre la volonté de créer de nouvelles places de prison, lesquelles ne seront disponibles que dans huit à dix ans, et la fermeture immédiate de places de bonne qualité actuellement disponibles à Clairvaux, alors même que nous connaissons tous le scandale de la surpopulation carcérale. Depuis l'annonce de la décision du ministère de la justice, la population s'est mobilisée

Nous sommes scandalisés par cette attitude, qui marque la volonté de rendre irrémédiable une décision tout à fait inacceptable, alors même que les différents candidats à l'élection présidentielle nous ont fait part de leur intention d'en suspendre l'exécution.

Failles de sécurité, isolement géographique, difficultés d'accès aux soins, coûts de fonctionnement et de rénovation exorbitants : tous ces éléments ont conduit à cette décision logique. J'ajoute que les maisons centrales, à ne pas confondre avec les maisons d'arrêt, qui sont en effet surpeuplées, ont un taux d'occupation de 76 % seulement, d'où la décision de fermer les établissements les plus coûteux, qui sont souvent aussi les plus vétustes.

Je vous indique que les agents qui le souhaiteront pourront être affectés dans tous les établissements de France métropolitaine, dans la limite d'un sureffectif de 15 %. Ils bénéficieront, en vertu d'un décret de 2009, d'une prime de restructuration allant de 12 000 à 15 000 euros. Pour coordonner la reconversion du site et le reclassement des personnels dans d'autres établissements pénitentiaires, un sous-préfet a été nommé le 4 octobre dernier. Trois missions lui sont confiées : atténuer les incidences de la fermeture de

La séance est reprise. Par lettre en date du 14 février 2017, M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître, conformément à loi organique n° 2010-2837 du 23 juillet 2010 et en application de l'article L.O. 567-9 du code électoral, l'avis de la commission des lois sur le projet de nomination, par M. le Président de la République, du président de la commission prévue au dernier alinéa

des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en oeuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé évoquer le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l'article 166

ont abouti à un accord sur les dispositions restant en discussion des projets de loi relatifs à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé- l'ANSM S'agissant du texte portant simplification de procédures mises en oeuvre par l'ANSM et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé, plusieurs articles restaient en discussion. L'article 2, relatif à l'obligation de déclarer les quantités de médicaments exportés, avait été substantiellement modifié par l'Assemblée nationale pour étendre cette obligation à tous les acteurs du système, et non aux seuls grossistes-répartiteurs. À la lumière des débats qui ont eu lieu au Sénat, cette position nous a paru pouvoir être suivie. L'article 3 tend à transposer une directive relative à l'importation de tissus et de cellules. Nous avons poursuivi en CMP l'important travail de coordination mené par nos deux assemblées.

Elle répondait à l'une des préconisations du rapport de notre commission sur la politique vaccinale. La CMP a entériné les précisions rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'adopter ses conclusions, qui ne font guère débat.

L'article 1, tendant à ratifier l'ordonnance créant Santé publique France, avait été adopté conforme. Notre assemblée a toujours été très favorable à la rationalisation du fonctionnement des agences sanitaires et des multiples organismes créés au fil du temps. C'est pourquoi elle a d'emblée soutenu la création de l'ANSP, issue de la fusion de trois agences préexistantes. La commission des affaires sociales avait néanmoins émis une réserve quant à la méthode employée par le Gouvernement. avant même sa ratification, le texte de l'ordonnance a été modifié par la loi de finances pour 2017. Celle-ci supprime le principe d'un financement de l'agence par l'assurance maladie. Cette instabilité est préjudiciable tant à la sincérité de nos débats qu'à la prévisibilité dont l'agence doit pouvoir bénéficier au moment où elle se met en place. L'article 2 du projet de loi restait pour sa part en discussion. Il s'agissait de modifier l'article 166 de la loi santé afin d'inclure l'ANSP dans le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement pour « adapter les dispositions législatives » en vue de la mutualisation des fonctions dites « support » de plusieurs organismes. Nous avons étudié la proposition du Gouvernement sans, en

Nous n'avons pas obtenu les précisions attendues. En quoi les dispositions législatives actuelles font-elles obstacle à des projets de mutualisation ? Quels sont les projets Quels sont les projets envisagés ? À ces questions simples, les réponses de nos différents interlocuteurs ont été évasives, changeantes, voire contradictoires. Nous ne sommes pas opposés par principe aux habilitations et aux ordonnances. Il faut toutefois pouvoir justifier d'une véritable nécessité juridique et faire preuve d'un minimum de transparence à l'égard du Parlement. C'est pourquoi le Sénat a supprimé cette habilitation

Il me paraît curieux, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement ne tienne pas compte des débats parlementaires en cours ... Certes, le texte de l'ordonnance, désormais publié, est différent du projet qui nous avait été transmis initialement. Peut-être nos remarques n'étaient-elles pas si infondées et ont-elles suscité certaines interrogations ? Néanmoins, il s'avère que le texte définitif, lui non plus, n'a pas véritablement pour objet d'apporter aux dispositions législatives en vigueur des modifications destinées à faciliter à faciliter les mutualisations. Il s'agit purement et simplement d'opérer un transfert définitif de compétence du pouvoir législatif au pouvoir réglementaire. Dans ces conditions, le projet de loi qui devra être déposé pour ratifier l'ordonnance ne pourra pas, de notre point de vue, être adopté en l'état sur ce point. Il ne me paraîtrait d'ailleurs pas infondé qu'une initiative parlementaire soit prise pour, éventuellement, supprimer les dispositions en cause.

nous nous retrouvons ce soir pour examiner, une dernière fois, deux projets de loi de ratification d'ordonnances issues de la loi de modernisation de notre système de santé, dont le processus législatif, entamé à l'automne, arrive à son terme. En effet, lors de la réunion du 17 janvier dernier, les deux commissions mixtes paritaires sont parvenues à des accords, d'une part sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en oeuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé, d'autre part sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique. Les deux textes proposés par la CMP ont été adoptés par l'Assemblée nationale le jeudi 26 janvier dernier, et c'est aujourd'hui au Sénat qu'il revient d'approuver- ou non -le travail de la commission mixte paritaire. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence nationale de santé publique. Vous le savez, l'ANSP réunit aujourd'hui l'Institut de veille sanitaire- l'InVS -, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé- l'INPES -et l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires- l'EPRUS. Quelques mois seulement après sa création, cette agence est pleinement intégrée dans le paysage sanitaire français. à cette ordonnance, l'Agence nationale de santé publique peut désormais intervenir dans l'ensemble du champ de la santé publique, de la production de connaissances à la préparation face aux menaces et à la gestion de crise sanitaire. Elle est également pleinement compétente pour élaborer des réponses efficaces dans le vaste champ de la promotion de la santé et de la prévention. L'épidémie de grippe que notre pays a traversée cet hiver a pu démontrer au plus grand nombre l'intérêt de l'action d'un opérateur de l'État qui, tout à la fois, surveille la dynamique de l'épidémie, fournit des données sur les populations ou les territoires les plus touchés et, en cohérence, propose au Gouvernement des mesures d'information des professionnels et de communication en direction du grand public. C'est la raison C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a soutenu la volonté des rapporteurs d'associer plus étroitement la représentation nationale à la définition des politiques de santé publique, en lui attribuant des sièges au sein du conseil d'administration de l'ANSP.

le Sénat en première lecture. La loi de modernisation de notre système de santé avait accordé au Gouvernement, dans les conditions précises fixées par l'article 38 de la Constitution, la possibilité de prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, toutes mesures législatives destinées à favoriser la mutualisation des fonctions transversales d'appui et de soutien entre les agences relevant des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

J'en viens au projet de loi de ratification de l'ordonnance portant simplification des procédures mises en oeuvre par l'ANSM.

Je ne reviendrai pas dans le détail sur ses apports. Au-delà des aspects techniques, il permet de moderniser en profondeur nos procédures de sécurité sanitaire, de compléter notre arsenal de lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments et de renforcer la gouvernance de la politique vaccinale. Je m'arrêterai néanmoins sur l'article 2, qui vise à expérimenter, pour les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, mais aussi pour les industries pharmaceutiques, la déclaration des quantités de médicaments produits ou acquis, non consommés au sein du système de santé français et exportés. Je me souviens évidemment très bien des débats que nous avions eus lors de l'examen de cet article devant votre commission et des interventions des sénateurs et sénatrices qui avaient alors relayé les inquiétudes des professions concernées. C'est pourquoi je suis heureuse que le travail effectué au cours de la navette parlementaire ait permis de rassurer les grossistes-répartiteurs, qui avaient pu se sentir injustement ciblés par cette expérimentation,

sera désigné en concertation avec tous les acteurs concernés. Cette mesure complétera utilement l'action engagée par Marisol Touraine pour lutter contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments, en renforçant la transparence et en donnant aux pouvoirs publics une meilleure visibilité sur les niveaux et contenus des stocks. Je conclurai en indiquant que le Gouvernement se félicite du large consensus- malgré quelques différends mineurs -ayant accompagné le processus de ratification de ces ordonnances et permis leur adoption dans un délai rapide. En soutenant ainsi la mise en place de l'Agence nationale de santé publique et la simplification des procédures de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la représentation nationale aura démontré, une fois de plus, son attachement unanime aux maillons essentiels de la politique de santé que constituent nos agences sanitaires. La parole est Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la loi santé prévoyait un grand nombre d'habilitations du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Je les avais accueillies avec une grande réserve. Mes collègues corapporteurs et moi-même avions proposé d'en supprimer plusieurs, compte tenu de la sensibilité des sujets concernés et de la difficulté à évaluer les conséquences des modifications affichées. Dans une démocratie, le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement ; il est le plein détenteur du pouvoir législatif. Le Sénat était donc dans son rôle, me semblait-il, en procédant de la sorte.

au fonctionnement et aux ressources de l'InVS, de l'INPES et de l'EPRUS, ainsi que de la future Agence nationale de santé publique, dans la mesure où ces agences étaient déjà concernées par une habilitation.

En première lecture, j'avais affiché ma prudence sur le projet de loi de ratification relatif à la création de l'agence nationale Santé publique France, au motif que le Gouvernement tentait d'utiliser cette habilitation pour opérer un transfert définitif

Le Parlement ne doit pas céder face aux tentatives des gouvernements, quels qu'ils soient, visant à circonscrire notre action. Je voterai, comme mon groupe, ce projet de loi délesté de l'habilitation portant sur les mutualisations.

L'expérimentation proposée ici est à saluer. Elle vise à s'assurer du volume globalement exporté, pour mieux appréhender les causes des crises. À l'origine, l'obligation de déclaration s'imposait seulement aux grossistes-répartiteurs. J'étais, en première lecture, favorable à ce que l'ensemble des maillons de la chaîne du médicament participent à cette expérimentation : les laboratoires, les distributeurs ou encore les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché. L'Assemblée nationale a ainsi élargi le champ de cette obligation de déclaration ; je m'en réjouis. Espérons que la communication de ces informations par tous les acteurs de la chaîne du médicament permette de comprendre l'origine des ruptures d'approvisionnement, afin que les solutions les plus adéquates

à condition, bien entendu, que les moyens financiers et humains ne soient pas diminués. Cela nous semble une évidence, et il serait souhaitable que celle-ci soit partagée par tous ...

le texte de l'ordonnance prévoit que la responsabilité du ministre de la santé soit transférée au directeur de l'ANSM, notamment en matière de détermination des bonnes pratiques de pharmacovigilance.

la simplification n'empêche pas les interrogations ! L'article 2 est, quant à lui, sociologiquement et philosophiquement intéressant. En effet, comment expliquer que, dans une société libérale marchande dont le commerce est presque devenu un des piliers, nous puissions

L'article 3 prête à discussion. En effet, certains d'entre nous sont, par principe, très opposés à la pratique d'une certaine marchandisation du corps humain et, en particulier, à l'importation de tissus ou de cellules humains en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne,

et prévoit des cadres pour l'importation et l'exportation de ces tissus. Mais le processus et la philosophie demeurent inchangés. À titre personnel, je dirais que ce qui est validé dans cet article 3 est logique et normal,

Heureusement, l'éthique existe encore. Mais, nous le savons très bien, l'histoire a montré que, dans le domaine scientifique, en particulier, l'éthique est parfois un peu élastique

Enfin, l'article 4 tend à organiser le transfert du Comité technique des vaccinations à la Haute Autorité de santé, afin de regrouper au sein d'une même instance ceux qui élaborent des recommandations vaccinales et ceux qui évaluent le service médical rendu. Cela nous paraît une très bonne chose. À propos des vaccins, permettez-nous permettez-nous de rappeler qu'il faut impérativement redonner à nos concitoyens confiance dans la démarche de vaccination et répondre, une bonne fois pour toutes, aux interrogations concernant les adjuvants, l'aluminium en particulier.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes réunis pour voter deux projets de loi visant à ratifier des ordonnances prises en application de l'article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé, les commissions mixtes paritaires ayant abouti à un accord sur ces deux textes le 17 janvier dernier. Je souhaite tout d'abord évoquer le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l'article 166 de la loi du 26 janvier 2016.

manque de cohérence et de lisibilité, les différents établissements ayant été créés en réaction à des crises, souvent sans cohérence d'ensemble. La nouvelle agence doit intervenir sur l'ensemble du champ de la santé publique, de la production des connaissances jusqu'à la gestion des crises sanitaires. Il s'agit de mieux connaître l'état de santé des populations, de comprendre ses déterminants et d'observer les signaux épidémiologiques, ainsi que d'assurer une veille sur les risques sanitaires. doit s'emparer de nombreux sujets : lutte contre le tabac, questions de nutrition ou encore inégalités de santé. La prévention est l'une de ses compétences les plus visibles, comme en témoigne la récente campagne « Moi(s) sans tabac ».

qui vise à assurer la représentation du Parlement au conseil d'administration de l'agence, aux côtés de représentants de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité et de l'Assemblée des départements de France.

et républicain du Sénat votera donc en faveur de l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence nationale de santé publique. texte élaboré par la commission mixte paritaire pour le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en oeuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé

L'article 2 de ce projet de loi prévoyait initialement l'expérimentation, pour une durée de trois ans, d'une obligation déclarative pour les seuls grossistes-répartiteurs concernant les médicaments qu'ils exportent. Les travaux de l'Assemblée nationale ont permis d'étendre cette expérimentation à tous les maillons de la chaîne du médicament, depuis la production jusqu'à l'approvisionnement. L'expérimentation concerne désormais les laboratoires pharmaceutiques, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, ainsi que les distributeurs en gros à l'exportation. Tous ces acteurs devront déclarer à un tiers de confiance les quantités de médicaments qu'ils exportent, dans le respect, bien évidemment, des exigences de confidentialité. Les sénateurs socialistes soutiennent cette mesure, car sa mise en oeuvre permettra de mieux estimer, en temps réel, les quantités de médicaments effectivement présentes sur le territoire français et d'apprécier la fluidité de la chaîne d'approvisionnement. Félicitons-nous que nos deux assemblées aient trouvé un accord sur ce point très important l'adoption d'amendements de coordination ou rédactionnels. tend également à transposer, au travers de son article 3, la directive européenne du 8 avril 2015 sur les procédures de vérification des normes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés. Cette directive encadre les conditions de l'importation, par les États membres de l'Union européenne, de tissus et cellules en provenance des pays tiers. Le rapporteur du texte au Sénat avait fait adopter en commission lors de la première lecture, avec l'accord du Gouvernement, tendant à rejeter toute possibilité d'importation directe de tissus et cellules depuis les pays de l'Union européenne et à imposer le passage par les banques de tissus et cellules contrôlées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Notre collègue Hervé Poher vient de rappeler les règles fondamentales d'éthique. Le projet de loi prévoit également, à la suite de l'adoption d'un amendement gouvernemental en commission des affaires sociales en première lecture, le transfert du Comité technique des vaccinations à la Haute Autorité de santé.

La création de l'Agence nationale de santé publique répond très largement à un souci de simplification et de rationalisation de nos politiques publiques. En effet, trois agences sont fusionnées, à savoir l'Institut de veille sanitaire, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et l'Établissement de préparation et de réponse aux et l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, pour former l'agence Santé publique France. Un sujet en particulier a fait l'objet de discussions avec le Gouvernement, au Sénat, et avec nos collègues députés en commission mixte paritaire : celui de l'habilitation donnée au Gouvernement de procéder par voie d'ordonnances à des modifications législatives aux fins de mutualisation de fonctions dites « support » de plusieurs organismes du champ sanitaire.

le Haut Conseil de la santé publique, l'Agence de la biomédecine ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mais l'inclusion de l'Agence nationale de santé publique dans le champ de cette nouvelle ordonnance nous semblait hâtive. Il eût été préférable que la fusion de l'InVS, de l'INPES et de l'EPRUS soit bien engagée avant de lancer une nouvelle mutualisation. C'est pourquoi la solution trouvée en commission mixte paritaire, consistant à ne pas inclure l'ANSP dans le champ de cette mutualisation,

L'article 2 de ce texte met en place une expérimentation, pour trois ans, visant à lutter contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments, que l'on ne compte plus depuis des mois. Initialement, le projet de loi limitait le champ de l'expérimentation aux seuls grossistes-répartiteurs. Il était pourtant nécessaire de l'étendre à tous les maillons de la chaîne du médicament, de la production jusqu'à l'approvisionnement. Je m'étais exprimée en ce sens en commission. mixte paritaire vise désormais les laboratoires pharmaceutiques, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et les distributeurs. L'ensemble de ces acteurs devront déclarer à un tiers de confiance, qui n'est pas défini dans le texte, les quantités de médicaments qu'ils exportent. La communication de ces informations doit permettre de comprendre l'origine des ruptures d'approvisionnement en médicaments. La mise en place d'un tel système risque d'être complexe. J'espère néanmoins que ce dispositif améliorera les analyses sur les exportations parallèles et leur lien éventuel avec les ruptures

Leurs causes sont nombreuses et multifactorielles. Il est urgent d'agir pour que les patients ne soient pas pénalisés. Par ailleurs, les autres dispositions de ce projet de loi, relatives par exemple à la transposition de la directive relative aux procédures de vérification des normes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés à des fins thérapeutiques ou au transfert des compétences du Comité technique des vaccinations à la HAS, n'appellent pas, de notre part, de remarques particulières. On l'aura compris, rien ne s'oppose à ce que le groupe Les Républicains approuve les conclusions des

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en préambule, je souhaiterais rappeler que nous ne sommes pas favorables à l'utilisation par le Sénat de la procédure d'examen en commission, dite

Concernant l'ordonnance relative à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dont l'objectif principal était la transposition d'une directive européenne relative à la qualité et à la sécurité des tissus et des cellules importés en provenance de pays tiers à l'Union européenne, notre groupe avait exprimé de nombreuses réserves lors de la première lecture. Nous sommes favorables à un meilleur encadrement de la commercialisation des produits issus de pays tiers, mais nous persistons à penser que la marchandisation de tissus et de cellules d'origine extra-européenne devrait être interdite au nom de l'éthique. Les amendements de précision introduits par l'Assemblée nationale ne lèvent pas totalement les risques potentiels de remise en cause, à terme, de notre modèle transfusionnel éthique, gratuit et bénévole. Pour ce qui est de l'expérimentation destinée à lutter contre les ruptures d'approvisionnement des pharmacies, nous nous réjouissons de l'évolution du texte, qui vise désormais non plus uniquement les grossistes-répartiteurs, mais aussi les laboratoires. Nous espérons que l'obligation de déclaration, pour les grossistes-répartiteurs, des quantités de médicaments qu'ils exportent

santé de rendre disponibles les trois vaccins obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. J'avais déjà eu l'occasion de dénoncer le fait que ces vaccins soient désormais associés à d'autres vaccins polyvalents, non obligatoires. Les industriels qui avaient organisé une rupture d'approvisionnement en arrêtant la production du vaccin DT-polio non associé à d'autres en 2008 seront donc, je l'espère, obligés de commercialiser de nouveau ce vaccin. Je serai, pour ma part, très attentive à ce que la décision du Conseil d'État soit bien suivie d'effet d'effet et que les trois vaccins obligatoires soient de nouveau disponibles et commercialisés. Il revient à Mme Touraine, ministre de la santé, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de ces vaccins. J'ajoute qu'il serait bon de mettre sur le marché des vaccins sans adjuvants aluminiques. Permettez-moi d'évoquer quelques-unes des mesures possibles. D'abord, la ministre de la santé peut sanctionner les laboratoires et les entreprises ne respectant pas « leur obligation d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion des pénuries de vaccins ». Elle peut également soumettre le brevet d'un médicament au régime de la licence d'office afin d'assurer sa mise à disposition en quantité suffisante. Enfin, elle peut saisir l'Agence nationale de santé publique, qui a le pouvoir de procéder à l'acquisition, à la fabrication, à l'importation et à la distribution de médicaments pour pallier une commercialisation ou une production insuffisante. Ces trois pistes de réflexion vont dans le sens de notre proposition

Il est donc indispensable que notre pays puisse disposer d'un établissement assurant une expertise globale, afin de garantir la protection sanitaire de la population. J'insisterai une nouvelle fois sur la question des moyens humains et financiers alloués à l'ANSP.

Nous avons le recul nécessaire pour constater que les politiques de santé menées depuis de nombreuses années vont à l'encontre des missions de service public. De toutes parts s'élèvent des voix appelant à modifier les choix qui sont faits. La souffrance au travail des personnels de santé n'est plus à démontrer, et plutôt que de vouloir gérer ce que l'on appelle pudiquement les risques psychosociaux,

un an après la promulgation de la loi de modernisation de notre système de santé, nous sommes appelés à nous prononcer sur deux projets de loi visant à ratifier des ordonnances. Sur ces deux textes, l'Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord. Le premier texte prévoit notamment la ratification d'une ordonnance portant création de l'Agence nationale de santé publique, appelée Santé publique France. La fusion de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est une très bonne chose.

Cette fusion permettra à la France de se doter d'un établissement d'excellence dédié à la prévention et à la promotion de la santé, à la veille sanitaire, à la surveillance et à la réponse aux crises sanitaires, à l'image des agences de santé américaine, anglaise et canadienne. À l'issue de la première lecture, seul un article restait en discussion : l'article 2, qui incluait l'Agence nationale de santé publique dans le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement afin d'adapter les dispositions juridiques en vue de favoriser ou de permettre la mutualisation des fonctions dites « support » de plusieurs organismes. Comme l'avait relevé en première lecture notre excellent rapporteur, Gilbert Barbier, « il apparaît que le projet d'ordonnance du Gouvernement n'a pas véritablement pour objet d'apporter aux dispositions juridiques en vigueur des modifications destinées à faciliter les mutualisations. Il s'agirait purement et simplement de renvoyer à un décret, voire à un arrêté, la mise en oeuvre de ces mutualisations et d'opérer ainsi un transfert définitif de compétences du pouvoir législatif au pouvoir réglementaire. L'étude d'impact est d'ailleurs très claire sur ce point : elle précise en effet que « les mesures envisagées aux I et II de l'article 2 du présent projet de loi auront pour conséquence d'élargir le champ des ordonnances prises sur le fondement des habilitations prévues prévues au 1° du III et au 1° du V de l'article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé ». Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire ait suivi la position de la Haute Assemblée.

est une sage décision, qui permettra au Parlement de garder toute sa compétence. La seconde ordonnance soumise à ratification simplifie les procédures mises en oeuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et comporte diverses dispositions relatives aux produits de santé. Je ne m'étendrai pas sur l'article 1, adopté conforme par les deux assemblées, qui simplifie les procédures de l'ANSM en vue d'alléger la charge de travail administratif pesant sur elle. Nous y souscrivons pleinement. Vous l'avez rappelé devant l'Assemblée nationale, madame la secrétaire d'État, l'ANSM est « un acteur central et indispensable de la surveillance des produits de santé et, plus généralement, de la sécurité sanitaire dans notre pays ». Ces mesures « permettront d'accompagner son évolution tout en garantissant à nos concitoyens le niveau de sécurité et de confiance qu'ils attendent s'agissant des produits de santé À l'issue de la première lecture, trois des cinq articles restaient en discussion, dont l'article 2, qui imposait initialement aux grossistes-répartiteurs, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de déclarer auprès d'un tiers de confiance les volumes de médicaments exportés.

Seront donc également concernés les laboratoires pharmaceutiques, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et les distributeurs en gros à l'exportation. Cette nouvelle rédaction permettra enfin d'assurer une traçabilité complète des médicaments présents sur le marché français et de lutter contre les ruptures d'approvisionnement, devenues devenues de plus en plus fréquentes ces dernières années : il s'agit d'un véritable enjeu de santé publique. L'Ordre national des pharmaciens a ainsi recensé près de 200 000 déclarations de rupture de stock entre les mois de février 2015 et de novembre 2016. Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe du RDSE suivront la position du rapporteur et approuveront ces deux textes. close. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, il se prononce par un seul vote

à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l'article 166 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.